le traitement des recettes de subventions dans le cadre de la période transitoire du prélèvement à la source. Un calcul sera fait en 2019 sur la base de la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019. Il en résulte que, pour 2019, les travaux ne sont pas déductibles en totalité, alors que les subventions qui contribuent à leur financement sont déclarées pour leur montant total en revenus. Cela s'avère d'autant plus inéquitable et contraire à l'esprit de la loi en cas de décalage dans le temps entre le paiement des travaux et la subvention, ce qui est malheureusement fréquent pour ce qui concerne les subventions d'État.

ne reportent de 2018 vers 2019 leurs dépenses de travaux et de permettre ainsi de préserver l'activité du bâtiment. Des règles spécifiques ont été prévues concernant la déductibilité des charges pour la détermination du revenu foncier net imposable au titre des années 2018 et 2019, en fonction de la nature de ces charges. Les charges récurrentes échues en 2018 sont admises en déduction au titre de cette même année, quelle que soit la date de paiement, et les charges pilotables de travaux sont admises en déduction en 2019 à hauteur de la moyenne des dépenses payées en 2018 et 2019 au titre de ces mêmes charges. C'est la règle de la moyenne, qui nous apparaît comme la plus équilibrée pour dissuader les contribuables de décaler leurs dépenses de travaux de 2018 sur 2019 et éviter une concentration des dépenses sur 2019. Ce faisant, nous considérons que cette mesure a permis de préserver l'activité du secteur du bâtiment en 2018.

La réforme n'aura par conséquent pas d'effet significatif sur l'activité du bâtiment considérée globalement, dont les moteurs sont la construction et les travaux réalisés dans les habitations principales ou secondaires. À nos yeux, la règle de la moyenne permettra de nous assurer que, même sur cette part très minoritaire de l'activité, l'impact de la réforme n'est pas significatif. Enfin, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de prévoir un traitement spécifique pour les dépenses payées à l'aide de subventions ou d'indemnités dans le cadre de la retenue à la source, dès lors qu'elles sont traitées à égalité avec les autres charges foncières déductibles. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut de l'année de leur encaissement par le bailleur et, corrélativement, les dépenses payées à l'aide de ces subventions ou indemnités sont déductibles des revenus fonciers. Dès lors, leur déductibilité dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source sera opérée selon le régime applicable en fonction de l'année de réalisation de la dépense. Ainsi, les dépenses payées en 2018 seront déductibles au titre des revenus de l'année 2018. S'agissant des dépenses de travaux payés en 2019, leur déductibilité sera égale à la moyenne de ces mêmes charges sur les années 2018 et 2019. Pour conclure, nous considérons que la mesure proposée conduirait à traiter plus favorablement des dépenses qui sont en partie subventionnées, et qui bénéficient donc déjà d'une aide publique. Nous ne saurions justifier une telle rupture d'égalité, au détriment des propriétaires qui ne reçoivent aucune subvention pour financer leurs travaux. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. La parole est à M. le rapporteur général.

parole est à M. Richard Yung. Cet amendement vise à apporter trois modifications au nouveau régime fiscal applicable aux revenus d'activité et de remplacement de source française perçus par les non-résidents. première modification concerne les abattements de 10 % dont il est actuellement fait application pour le calcul de la base de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Les nouvelles dispositions du code général des impôts précisent que les non-résidents ne pourront plus bénéficier ni de l'abattement pour frais professionnels ni de l'abattement en faveur des pensionnés et retraités. Nous proposons de rétablir ces deux de rétablir ces deux abattements. La deuxième modification concerne le taux minimum d'imposition. Le Gouvernement propose de faire passer ce taux de 20 % à 30 %. Quelle surprise désagréable

Nous proposons donc de maintenir le taux minimum d'imposition à son niveau actuel, c'est-à-dire à 20 %. La troisième modification concerne les charges que les non-résidents peuvent déduire de leurs revenus mondiaux

fin de son propos. Le relèvement du taux minimum n'aura d'impact que pour les contribuables dont le taux moyen d'imposition sur les revenus mondiaux est supérieur à 20 % ; la situation des contribuables dont le taux moyen est déjà inférieur à 20 % n'est pas modifiée. Par ailleurs, il faut souligner que cette mesure incitera les contribuables à déclarer plus systématiquement leurs revenus mondiaux afin de bénéficier du taux moyen, conformément aux recommandations du rapport sur la mobilité internationale des Français remis par la députée Anne Genetet. Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

qui fait de vous la première puissance géostratégique du monde, qui vous permet, en bombant le torse, de dire : « Jamais le soleil ne se couche en France ! » Pourtant,

qui est en voie de développement, en tout petit, petit, petit développement, il fallait s'attaquer aux classes moyennes, en particulier à la tranche basse de la classe moyenne. Cette théorie économique ne tient pas la route.

que nos compatriotes ne se sentent pas méprisés et stigmatisés quand, sourds à nos remarques et aveugles à nos réalités, vous insistez sur le bien-fondé de mesures fiscales que nous nous évertuons à décrire comme dangereuses pour nos économies et complètement iniques

où est l'équité quand, par un tour de passe-passe budgétaire, vous augmentez l'impôt pour 20 % des citoyens ultramarins, à hauteur de 10 % au minimum- cette mesure impactera également le monde de l'entreprise les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux -, augmentation couplée, pour certains, avec celle de la CSG Où est l'équité quand on demande aux régions d'outre-mer de participer seules au financement des investissements publics et à la moitié des territoires ultramarins, des DOM pour être précis, pourtant déjà dans une situation économique délicate, voire critique, de participer seuls au financement de dispositifs situés aussi dans les COM, où l'impôt sur le revenu n'est pas applicable ? Sur quel territoire de France continentale cela s'est-il déjà vu ? Vous donnez l'impression que nos citoyens sont des enfants gâtés. Il n'en est rien, monsieur le secrétaire d'État ! L'abattement supplémentaire de l'impôt sur le revenu compense la cherté de la vie et la rupture d'égalité qu'entraînent l'éloignement et l'insularité de nos outre-mer. Je m'oppose farouchement à ce nouveau coup de rabot d'au moins 70 millions d'euros censé alimenter un fonds dont nous ne connaissons ni la répartition ni l'efficacité. Sur la base de motifs fallacieux,

le Gouvernement ayant présenté sans discussion aucune et de manière fort unilatérale une mesure qui consiste, au nom de la lutte contre les inégalités, à faire

d'environ 1 000 euros par dossier fiscal, est-il forcément la meilleure entrée pour poser la question du développement de nos outre-mer ? C'est une question récurrente, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans cette enceinte. Je rappellerai qu'il ne s'agit sans doute coup, de la principale dépense fiscale à l'oeuvre dans ces territoires de la France du monde entier et que la critique d'efficacité adressée à la réduction générale de l'impôt ne saurait lui être réservée. Les modes de défiscalisation des investissements en vigueur,

si l'on en croit l'évaluation des voies et moyens et le « bleu » de la mission « Outre-mer », les dépenses fiscales associées devraient s'élever, en 2019, à plus de 4,6 milliards d'euros, dont 1,9 milliard d'euros correspondant aux effets du moindre taux de TVA applicable aux livraisons de biens et de services dans les DOM et près de 1,3 milliard d'euros liés à la non-application de la TICPE. On sait que cette dernière est remplacée par une taxe propre aux DOM, dont le rendement s'avère au demeurant assez proche des sommes non perçues au titre de la TICPE. Autant dire que les 110 millions d'euros que l'État escompte récupérer avec les mesures de cet article 4 ne vont qu'assez peu entamer les dépenses fiscales existantes. La question qui demeure toutefois posée, s'agissant de l'article 4, est connue : oui ou non la vie est-elle chère dans les DOM, compte tenu des règles de sujétion commerciale imposées par la métropole à ces territoires ? Si elle est chère, ce que semble montrer avec éclat le niveau actuel de la mobilisation populaire dans l'île de La Réunion, par exemple, est-ce le meilleur moment pour rectifier une mesure dont l'un des fondements était précisément de lutter contre la vie chère ? Nous ne le pensons pas ! Il nous semble même que les tensions toujours vives que connaissent d'autres territoires d'outre-mer, pour des raisons diverses- je pense à Mayotte ou à la Guyane -, appellent une réflexion plus complète et plus concrète sur la situation de ces Français du monde entier que sont nos compatriotes ultramarins. C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l'article 4. La parole est à M.

utilisées pour abonder le budget des outre-mer. Notre volonté est vraiment de flécher ces recettes ; Annick Girardin, ministre des outre-mer, l'aurait dit devant vous si elle n'avait pas dû rejoindre l'île de La Réunion pour

pour l'ensemble des ministères, un investissement total de 2,1 milliards d'euros dans les futurs contrats de convergence et de transformation. Par exemple, 50 % de l'enveloppe nationale qui sera dédiée en 2019 aux investissements hospitaliers sera consacrée aux hôpitaux ultramarins. De la même manière, nous augmentons de près de 300 millions d'euros, pour 2019, les crédits consacrés à l'outre-mer sur l'ensemble des périmètres interministériels. Nous veillons à travailler avec l'ensemble des outre-mer, et il faut souligner que les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu que nous présentons

en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, une famille avec trois enfants ne sera concernée qu'au-delà de 96 000 euros de revenus annuels. Un professeur du secondaire à La Réunion ne verra son impôt augmenter que de 4 euros par mois.

laquelle la solidarité ultramarine doit jouer avant la solidarité nationale. Soit ! Mais ne nous trompez pas avec des chiffres qui sont absolument faux. Ne nous dites pas

note dans laquelle on a trouvé tellement d'incohérences, tellement de contre-vérités, tellement de contresens que Mme la ministre a finalement dû consentir, avant son départ à La Réunion, hier matin, à nous recevoir

c'est qu'on nous avait vendu ça ( un suivi transparent, 1 milliard d'euros fléchés pour les outre-mer dans le grand plan d'investissement, un compteur public qui afficherait sa réalisation ! Et que nous dit-on

et déclarant plus de 92 000 euros annuels ou encore, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, une famille de trois enfants, avec plus de 96 000 euros de revenus annuels. Troisièmement, vous me pardonnerez de le dire brutalement, il est compliqué- la ministre de l'outre-mer vous l'aurait dit comme moi -d'entendre dire qu'il y a une absence de solidarité quand, comme je l'ai rappelé, 2,1 milliards d'euros seront investis dans les plans de convergence, quand 50 % de l'enveloppe des investissements hospitaliers sera consacrée aux outre-mer, quand nous augmentons le périmètre budgétaire des outre-mer de 300 millions d'euros en 2019. ! Il est tout aussi difficile, monsieur Lurel, de pointer l'absence de solidarité quand l'effort budgétaire de l'État par habitant est supérieur de 50 % à celui de l'Hexagone ou quand les taux de prélèvement y sont plus de 10 points inférieurs, faisant des départements et régions d'outre-mer des territoires où le niveau de taxation est à peu près équivalent à celui des pays les moins taxés de l'Union européenne, comme l'Irlande ou la Lituanie. Cela fait partie des éléments qui nous amènent à ne pas être d'accord, je le

d'un amendement de repli, car il ne nous reste plus que ça : nous replier derrière notre misère, nous replier derrière notre sous-développement, nous replier derrière la sous-considération,

À titre liminaire, je ne peux m'empêcher de m'étonner du procédé sans précédent qui consiste à augmenter dans de telles proportions les impôts outre-mer pour y financer par ailleurs des mesures. financer par ailleurs des mesures. Je le dis comme je le pense, ce procédé et la réduction de l'abattement qui en découle me semblent économiquement absurdes ! Même si l'on admet que la réduction de l'abattement ne concerne que les catégories supérieures, il n'en reste pas moins que, macroéconomiquement, il s'agit d'une augmentation d'impôt. Elle sera de 1 534 euros en moyenne, selon les chiffres du Gouvernement, montant qui n'a pas la même résonance selon l'endroit où l'on se situe sur l'échelle des catégories dites « supérieures Dès lors, dans tous les cas, cette augmentation d'impôt se traduira immanquablement par une baisse de la consommation, dont les effets ne seront pas nécessairement compensés par les dépenses au titre du FEI puisqu'elles stimuleront l'investissement et non la consommation. Nous ne devons pas non plus occulter l'impact psychologique de la réduction de l'abattement. Interprétée comme l'annonce de sa suppression définitive à plus ou moins court terme, elle engendrera un comportement de prudence ou de méfiance, y compris de la part des contribuables qui ne sont pas concernés. une réduction de la consommation, qui pourrait se traduire par une augmentation de l'épargne de prudence. Enfin, replacée dans le contexte de la politique budgétaire outre-mer pour 2019, la réduction de l'abattement devient un facteur supplémentaire du climat récessif qui s'annonce sous l'effet des mesures cumulées.

Cet étalement offre de surcroît le mérite d'évaluer les effets du dispositif au bout d'un an.

L'investissement de l'État est de 10 000 euros moins élevé dans l'outre-mer qu'en France ! Où a-t-il pris ces chiffres ? L'INSEE est un institut national

au ministère des outre-mer, parce qu'il fallait tout revoir et tout recommencer ? Même les socio-professionnels de nos pays n'ont pas accepté la farine dans laquelle nous étions roulés

tous les voies et moyens, de trouver une manière de compenser un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, en particulier pendant les campagnes électorales,

exactement comme lors de la crise guyanaise, le tout sans avoir à aucun moment les moyens de financer les retards de développement qui ont été pris. Eh bien, assumez, et on verra ! Rendez-vous dans trois ans et demi

il est important que nous participions, dans les temps qui sont les nôtres, à l'effort national. Mais lorsque l'effort est plus que difficilement

Il me vient à l'esprit, et mon collègue Lurel s'en rappellera très certainement, ce fameux livre qui a fait couler tant d'encre :. Comme si nous étions une charge et uniquement une charge pour la France

les règles de fiscalité qui s'appliquent aux pensions de source française versées dans les collectivités d'outre-mer historiques de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Compte tenu de la taille du territoire, les pensions servies à Saint-Barthélemy sont nécessairement considérées comme des revenus de source française en l'absence de possibilité d'établissement sur le territoire pour les organismes de retraite. Je rappelle que tous les revenus de source locale sont imposés localement. De plus, le dispositif que je vous propose doit être examiné en ayant en tête l'augmentation prévue par le présent texte de la fiscalité sur les non-résidents fiscaux de 20 % à 30 %. à 30 %. Cela peut paraître surprenant, mais un habitant de Saint-Barthélemy est considéré comme un Français de l'étranger ... Il convient d'en atténuer l'impact éventuel sur les pensionnés de ce territoire qui seraient soumis à l'impôt. C'est aussi une mesure de clarification de l'imposition à laquelle peuvent être soumis les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy. Tel n'est pas le cas en l'absence de convention fiscale. Pour être tout à fait précis, il s'agit d'une mesure de précaution dans la perspective de la mise en place du prélèvement à la source, bien qu'il ne s'applique pas en tant que tel aux non-résidents fiscaux, pourrait avoir un impact sur la fiscalité des pensions à Saint-Barthélemy. En outre, l'impact budgétaire de cette disposition est totalement négligeable : le dernier recensement du nombre de bénéficiaires d'une pension de retraite était d'environ 400 retraités. Enfin, Enfin, quant au risque d'appel d'air, et donc d'installation à Saint-Barthélemy de nouveaux retraités, il est là encore négligeable, pour au moins trois raisons. La première est la clause de cinq ans avant l'acquisition de la résidence fiscale, qui aggrave la deuxième raison, le coût de la vie. vie. La troisième tient à la taille du territoire : sur un territoire de 21 kilomètres carrés, il est impossible de disposer de l'ensemble des spécialités médicales, par exemple, ce qui constitue un frein à la mise en oeuvre du cliché de la retraite au soleil. Si l'on reste à Saint-Barthélemy une fois à la retraite, croyez-moi, on s'y installe rarement à ce moment de sa vie. Je crois donc que l'extension de cet abattement ne fait peser, pour ces raisons, aucun risque sur les finances de l'État.

Défavorable.

J'accepte de poursuivre la parodie de démocratie dans laquelle nous sommes. Oh là là ! On nous demande de voter des choses qui sont finalement déjà largement arrêtées, et il n'est pas question de bouger une virgule ou le moindre chiffre

Antiste, sur l'article. La TVA NPR est une particularité régionale que mes collègues ultramarins connaissent très bien. Ce dispositif constitue une aide indispensable à l'investissement

que ce mécanisme était inefficace, peu traçable, non piloté, avec des effets sur le développement économique illisibles. Où est l'étude d'impact nourrie et approfondie qui sous-tend cette déclaration Je considère, pour ma part, que le réajustement brutal de ce dispositif, sans en avoir une évaluation précise, risque surtout de déstabiliser certains secteurs économiques, comme le BTP, et le tissu économico-industriel, déjà en en souffrance. Ensuite, vous nous affirmez que la suppression de cette taxe sera complètement compensée par la création d'un dispositif de crédits d'intervention d'un montant de 100 millions d'euros par an. Comment le sanctuariserez-vous dans le temps ? Quels seront les outils plus efficients que vous nous promettez en contrepartie ? Quel est le calendrier de leur mise en oeuvre ? Autant de questions sans réponse qui montrent l'empressement du Gouvernement, incompatible avec les intérêts de nos territoires et de nos entreprises. De plus, la TVA NPR est utilisée aujourd'hui comme un outil de subvention à l'investissement pourvoyeur d'emplois, dans des territoires en effet très sinistrés à ce niveau. Ce dispositif, je le rappelle, présente l'avantage d'être directement mobilisable par les entreprises et simple dans son utilisation. Il n'est pas non plus soumis à une quelconque procédure d'agrément. Les outils mis en oeuvre ultérieurement auront-ils la même souplesse et la même efficacité ? Je crains que l'on n'aboutisse, ni plus ni moins, à une énième logique de subventionnement décidée par Paris. Enfin, le coût de ce dispositif était estimé à 224 millions d'euros avant 2009, puis à 100 millions d'euros ces dix dernières années, alors que vous avez indiqué à l'Assemblée nationale que ce montant n'était finalement que de 23 millions d'euros. Combien coûte-t-il réellement ? Le Gouvernement en a-t-il seulement une idée ? De sérieux doutes nous ont conduits à déposer un certain nombre d'amendements sur le sujet. La

dans la mission « Outre-mer », sont désormais gérées, comme vient de le dire Maurice Antiste, par le ministère, avec tous les problèmes d'exécution, de régulation de gel et de surgel

taxer la réserve des compagnies d'assurances s'il voulait réorienter l'épargne. Qu'est-ce que ce gouvernement et le Président de la République ont contre la liberté d'affecter librement son épargne ? Voilà l'une des raisons pour lesquelles

la majeure partie de la ressource ainsi mobilisée est un outil de financement du développement des entreprises ultramarines, alors même que nous ne sommes absolument pas certains de la qualité et la quotité des ressources que l'État va désormais consacrer à l'outre-mer. l'outre-mer. Les crédits de la mission en 2019- faut-il le rappeler ? -atteindraient 424 millions d'euros. Sur le montant total des crédits, 1 375 millions d'euros vont à l'allégement du coût du travail, en progression de 350 millions d'euros pour l'exercice 2018 ! En clair, les sommes récupérées sur la dépense fiscale, toujours largement orientées en direction des entreprises et des investisseurs, sont encore une fois mobilisées pour la version la moins pertinente de l'action publique. moins pertinente de l'action publique. Quand prendrez-vous enfin en compte la réalité des entreprises ultramarines ? Quand prendrez-vous en compte le fait que le secteur bancaire est insuffisamment mobilisé pour le développement économique local, d'autant que l'épargne des résidents est souvent captée par des investissements n'ayant aucun intérêt concret pour l'outre-mer ? En attendant, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l'article 5.

renforcée. La TVA NPR est une mesure de trésorerie dans un contexte d'accès au crédit, y compris à court terme, plus difficile qu'en métropole- il ne faut pas perdre cela de vue. Cela confère au mécanisme de TVA NPR un effet correctif qu'il convient de ne pas négliger. De plus, qu'on en qu'on en approuve ou non le principe, il n'en demeure pas moins que la TVA NPR est intégrée au calcul prévisionnel des entreprises auxquelles elle s'applique. Une remise en cause sur les produits qui devraient y être soumis constituerait donc un facteur déstabilisant pour la trésorerie de certaines entreprises. Ainsi, en fixant la date limite de livraison pour les biens commandés avant le 1 janvier 2019, et pour lesquels un acompte aura été versé au 1 juillet 2019, certains biens pourtant éligibles, puisque commandés en 2018, mais livrés en 2019 en raison des délais de fabrication, se retrouveraient exclus du dispositif. Je propose donc un aménagement de la disposition transitoire définie par le présent article, afin que la suppression du mécanisme de la TVA NPR ne produise pas d'effet pénalisant pour les commandes engagées en 2018. Cet amendement prévoit, par ailleurs, de limiter le bénéfice de la TVA NPR aux entreprises relevant des secteurs de compétitivité renforcée. Cette proposition procède de la conviction que, renforcer la compétitivité des entreprises ultramarines, suppose de ne pas s'arrêter au milieu du gué. Tous les moyens doivent donc leur être donnés, en tenant compte de l'écart des coûts de production avec leur environnement immédiat et de l'impossibilité pour les marchés exigus de réaliser des économies d'échelle. J'ajouterai un point qui n'a pas été

mer, qui vient grever le coût des marchandises entrant sur le territoire. L'aide à l'investissement était donc en partie, sinon totalement, justifiée.

une catastrophe pour les territoires ultramarins et porterait en l'état un coup sévère et brutal à des professions déjà sinistrées. Au motif de vouloir faire des économies, on s'attaque à des dispositifs pourtant nécessaires pour des territoires, exsangues, d'autant que cette mesure serait mise en oeuvre sans étude d'impact préalable quant à ses conséquences sur la santé économique et financière des départements d'outre-mer. Élus et acteurs économiques sont particulièrement inquiets du devenir de cette disposition, puisque la suppression de ce dispositif conduirait à la disparition d'une subvention de l'ordre de 8,5 % à peu près en Martinique et à La Réunion. Au regard de la situation économique et sociale de nos territoires, notamment en matière de chômage, et sans proposition alternative de nature à satisfaire les acteurs économiques et les élus, il est proposé d'introduire le report dans les DROM de la suppression de la disposition relative à la TVA non perçue récupérable, le temps que soient adoptés les plans de convergence prévus par la loi Égalité réelle outre-mer. Quel est l'avis de la commission

L'article 5 relatif à la suppression de la TVA NPR a été modifié par l'Assemblée nationale, afin de préserver de la suppression de ce dispositif les opérations engagées en 2018 pour lesquelles la livraison ou l'importation du bien intervient en 2019.

du bien fixée au 1 juillet 2019, ne couvrira donc pas le spectre de la plupart des biens concernés. Le présent amendement vise à décaler de six mois la date de livraison du bien par rapport au texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

M. Maurice Antiste. Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l'art en outre-mer, en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant, vivant, celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents, mais que leur pratique reste souvent celle d'amateurs. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d'autres territoires. Cet amendement a donc pour objet d'alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée.

de revenir à un dispositif de zonage qui ne soit pas géographique mais d'activité. Pour moi, c'est une mesure de bon sens, et j'ai envie de crier très fort : « Enfin ! » Enfin ! » Autrement dit, on ne peut pas considérer qu'un tiers, un dixième, un quinzième du territoire, sur un lieu précis, soit concerné par des mesures d'allégement, des mesures de compétitivité, et qu'on y

en mettant, d'un côté, des activités traditionnelles, comme le BTP, mais avec un dispositif de compétitivité renforcée, autrement dit avec un bonus particulier porté sur un certain nombre de mesures,

dans la Caraïbe. Il faut simplement veiller à ce que des mesures qui avaient été oubliées dans le zonage de compétitivité y soient aujourd'hui réintégrées. Dans son empressement, le Gouvernement a délaissé le transport régional. Comment pouvez-vous passer de la partie la plus importante de la Guadeloupe au reste de l'archipel si vous n'avez pas des moyens de transport aérien et maritime, avec les mesures de soutien qui vont avec ? peut-on considérer que la presse et tout ce qui touche au numérique ne soient pas concernés, alors que nous sommes sur des marchés contraints ? On sait très bien qu'un quotidien ou une télévision, dans ces pays-là, ne peut pas avoir les mêmes audiences, donc les mêmes recettes, qu'un média dans un pays disposant d'un marché, comme la France. Nous veillerons à ce que ces différentes ces différentes natures de secteurs soient préservées dans la mouture que nous allons voter au Sénat, autrement dit des secteurs à fort potentiel de développement.

et de ces zones la comptabilité, l'ingénierie, les études techniques et que sais-je encore ? Pourquoi avoir ôté la condition de financer la formation professionnelle pour en bénéficier ?

? Le régime des activités industrielles et artisanales dans ces zones franches est extrêmement coûteux.

Les taux d'exonération de l'imposition sur les bénéfices, de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties seront relevés dans tous les territoires et majorés en Guyane et à Mayotte, ainsi que dans les secteurs prioritaires exposés à la concurrence. Cette réforme est utile et attendue. Nous sommes donc défavorables à la suppression de l'article.

Cet amendement de repli vise à conserver cet article, en supprimant néanmoins les mesures qui paraissent injustifiées la remise en cause de la contribution à la formation professionnelle, qui conditionnait jusqu'alors le bénéfice des abattements fiscaux ; celle des dispositifs fiscaux majorés actuellement réservés à certaines zones géographiques,

de la réparation, de la transformation au dispositif d'abattements fiscaux majorés de la nouvelle zone franche d'activité nouvelle génération. En intégrant partiellement les activités industrielles, le dispositif actuel laisse de côté une part de ce secteur pourtant intégrée au dispositif de compétitivité renforcée en ce qui concerne des exonérations de cotisations patronales. Il serait cohérent d'intégrer l'ensemble des secteurs industriels, par symétrie et pour favoriser une synergie des deux mesures : exonérations et ZFANG. Je vous propose donc de tenir compte de l'ensemble des secteurs industriels sans restriction, pour favoriser la compétitivité de l'économie.

Territoire en forte croissance démographique, les moins de vingt ans sont majoritaires, mais leur scolarisation souffre d'un retard important par rapport à ceux de la métropole, et tant l'université que la formation professionnelle émergent à peine. c'est une île qui souffre d'un retard de développement économique : le PIB par habitant est 3,5 fois moins élevé que le taux national. Les entreprises ont encore besoin d'être accompagnées et soutenues pour se développer, se structurer et répondre à leurs obligations légales et réglementaires. Or si l'on veut y attirer les professions réglementées, les sociétés d'ingénierie et de conseil, il faut les intégrer au nouveau dispositif des ZFANG. Le Gouvernement, dans un contexte de budget contraint, fait certes

Les avantages fiscaux qui sont consentis à ces zones franches doivent évidemment permettre aux entreprises de lutter contre la concurrence. Ce sont donc des avantages qui sont normalement réservés

Monsieur le rapporteur

M. Maurice Antiste. J'ai soudain envie de soulager l'impatience de mes collègues, et je leur promets de ne pas

de « nuancer » le classement qui dépendait par trop de la densité des territoires, et de leur déclin, a introduit le critère du revenu fiscal des ménages. À cette occasion, elle a néanmoins surpondéré le système au profit du revenu fiscal par unité de consommation médian, qui intervient à parts égales et cumulativement au détriment des territoires faiblement peuplés et sans tenir compte de leur tendance à un déclin réel. Vous le savez, ce système a été prolongé jusqu'en 2020. Pour cette raison, une correction a été apportée, consistant en la réintroduction des EPCI en très fort déclin, à condition qu'ils se trouvent dans un arrondissement composé majoritairement de communes et d'une population classées en zone de revitalisation rurale. Il subsiste cependant le cas d'EPCI à très faible densité, telle qu'elle témoigne d'un déclin structurel, que le faible dépassement du revenu fiscal fait basculer en dehors du zonage par l'effet de la surpondération du deuxième critère. En réalité, on ne se sert que de deux critères

moins de 12 habitants au kilomètre carré et qui vient de sortir d'une ZRR au motif que sa population a un revenu médian supérieur de 0,6 % par rapport à la moyenne-

ont été proposés par deux de nos amis députés qui n'en ont peut-être pas mesuré complètement les effets, à moins qu'ils ne les aient trop bien mesurés ... J'estime qu'il faudrait se pencher très activement sur ce sujet, parce que ce sont des zones entières qui sont en train de perdre ces avantages pour des motifs complètement futiles. Lorsqu'on s'apercevra du déclin, il sera beaucoup trop tard. À l'heure actuelle,

Selon l'article 1465 A du code général des impôts sont en effet classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propre qui satisfait aux conditions énumérées par cet article, lesquelles portent sur la densité- faible -de la population et le revenu par habitant, qui doit être inférieur à un certain montant. Les zones de montagne sont définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, selon lequel ces zones « se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques ». On peut donc imaginer que, dans bien des cas, les communes situées en zone de montagne entrent, à leur échelle, dans les critères posés pour le classement en zone de revitalisation rurale. En revanche, la prise en compte de l'échelon intercommunal pour l'application de ces critères peut tout à fait entraîner une situation défavorable. Pour échapper à cet écueil, mon amendement vise à instaurer une exception, en prévoyant que, pour les communes situées en zone de montagne, mais appartenant à un EPCI dont le territoire n'est pas entièrement situé en zone de montagne, l'appréciation des critères de l'article 1465 A du CGI se fait au niveau communal. Quel est l'avis de la

des règles qui ont été posées récemment, nous préférons donner un avis défavorable ou demander le retrait de l'amendement afin de retravailler de manière plus globale ces questions, sachant que les communes, je le répète, sont protégées jusqu'en 2020.

prend en compte des intercommunalités qui ont une densité de population inférieure à 63 habitants au kilomètre carré. Ce qui pose problème, comme le souligne notre collègue, c'est le revenu médian par habitant, puisqu'il est situé autour de 19 100 euros.

car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements hyper ruraux. Déjà proposée l'an dernier, cette mesure de bon sens permettrait aux centralités des départements les plus éloignés de continuer de jouer leur rôle de locomotive économique et sociale du territoire et de donner une unité aux actions engagées par ces territoires pour développer leur attractivité d'une seule voix. Alors que se manifeste par de nombreux canaux la réalité de cette fracture entre la France connectée aux réseaux routier, ferroviaire, numérique et aérien et la France hyper rurale, dite « ruralité de l'éloignement », soutenir ces territoires éloignés et les initiatives qui s'y développent est essentiel. L'amendement n°

? Même avis. J'ajoute, y compris pour compléter la réponse apportée aux intervenants sur les amendements précédents, que le projet de loi

L'article 244 E du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt qui concerne les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition et réalisant certains investissements productifs en Corse, pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés- biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens et travaux de rénovation d'hôtel ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d'en bénéficier. Ce dispositif pourrait être élargi afin de bénéficier à l'ensemble des investissements des établissements de santé : construction, rénovation, investissements matériels et techniques.

cite, parmi la liste des biens qui peuvent déjà bénéficier de ce régime fiscal, les installations à caractère médico-social. Notre analyse, c'est que cela pourrait être déjà couvert

L'objet de cet amendement est de supprimer un article nouveau introduit par l'Assemblée nationale et qui vise à exclure les meublés de tourisme de l'éligibilité au crédit d'impôt sur les investissements en Corse, S'il a été constaté que le crédit d'impôt sur les investissements a été dévoyé pour l'acquisition de biens échappant ensuite au secteur touristique marchand et faisant office, dans les faits, de résidences secondaires, il faut évidemment y remédier, notamment par des contrôles accrus ou en l'assortissant d'une série de conditions qui pourraient par exemple être liées à un nombre minimal de logements, mais il ne faut pas le faire au détriment de projets professionnels réels. La citation expresse des meublés de tourisme, qui se trouveraient privés du bénéfice du crédit d'impôt, peut poser de sérieux problèmes dans une île où la création d'offres professionnelles est encouragée pour favoriser une économie réelle autour de l'activité Le CIIC actuellement en vigueur prendra fin le 31 décembre 2020. Dans la perspective d'une prorogation après cette date d'un dispositif toiletté, il serait préférable de supprimer cet article portant sur l'exclusion des meublés de tourisme et de mettre à profit les deux exercices qui nous restent pour trouver une rédaction appropriée, ne pénalisant pas les professionnels exerçant dans le cadre d'hébergements touristiques tels que les meublés de tourisme, tout en remédiant au dévoiement du dispositif. Quel est l'avis de

est déséquilibré le marché de l'immobilier, notamment des meublés, à l'échelle de la Corse. La suppression de ce secteur du champ des exonérations est donc une manière d'y répondre. Par conséquent, nous nous opposons à l'adoption de cet amendement.

ou TEOM- on dénombre plus de 2 000 affaires pendantes. Cet article sécurise les collectivités locales en élargissant le champ des dépenses prises en compte pour le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Néanmoins, il limite cet élargissement au programme de prévention des déchets ménagers ainsi qu'à la part incitative. Cet amendement vise

le Conseil d'État a évoqué un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses. L'amendement vise donc à définir ce taux en acceptant un écart de 15 % entre le produit de la taxe et les dépenses engagées pour ces missions. Cet ajout permettrait de définir plus précisément cette notion de disproportion limitée entre les recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût du service public de gestion des déchets. Pour information, cet amendement a été adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, mais il a ensuite été rejeté lors de son examen en séance.

public. Le Conseil d'État a rappelé que seule est admise une disproportion « limitée » entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd'hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse planer une incertitude pour les collectivités.

pouvant être prises en charge mais sans faire de lien avec le service public de gestion des déchets et sa comptabilité associée. Aussi, la seconde partie de l'amendement a pour objectif de clarifier opérationnellement les dépenses pouvant être couvertes par la TEOM.

de ces principes est que le montant de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport aux dépenses ; ce contrôle s'exerce par rapport aux dépenses prévisionnelles et non par rapport à l'exécution.

conduirait à inclure ni même de savoir si ce service relève de la compétence des collectivités en capacité d'instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par conséquent, nous craignons que l'élargissement

parfois, c'est dans une moindre mesure. Où est la bonne mesure ? Il porte là-dessus, le doute des contentieux, et c'est, à mon avis, ce qu'il faut purger. En revanche, vous vous posez la question d'inclure les frais de propreté de voirie

alinéas 4 à 8, qui précisent la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM. Cette disposition est contraire à la nature fiscale de la TEOM, qui est un impôt ; il n'y a donc pas lieu d'affecter les recettes aux dépenses. Ces dispositions rapprochent le régime de la TEOM de celui de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ce qui conduit à avoir deux types d'imposition pour le même objet.

Cet amendement vise donc à préciser la manière dont ces charges peuvent être intégrées, afin d'éviter de nouveaux contentieux. La l'amendement n° I-900. Il s'agit, au travers de cet amendement, d'utiliser un ratio pour sécuriser le rattachement des dépenses indirectes et des charges de structure dans le calcul des dépenses prises en compte pour la TEOM. est que ce ratio corresponde à la part des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets dans les dépenses globales. Cela permettrait d'avoir un ratio uniforme, objectif et facile à calculer, pour prendre en compte les frais indirects

l'amendement n° I-648. Cet amendement vise à clarifier les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.

: La parole est à M. Patrick Chaize. Le présent amendement a pour objet de dimensionner la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport à la réalité du service rendu, en prenant en compte les frais directs et indirects engagés par la collectivité. permettrait de clarifier la nature des charges prises en compte dans le calcul de la TEOM et de sécuriser l'action des collectivités locales. Il tend en outre à favoriser la mise en cohérence avec la comptabilité analytique prévue pour le service public de prévention et de gestion des déchets, dont la méthode de calcul retenue est une application concrète.

car les contentieux pèsent sur les contribuables. Il est à noter que la rédaction actuelle du projet de loi n'est pas applicable et fait peser de nouveaux risques de contentieux sur les collectivités, car le suivi dans la durée serait trop complexe. Il s'agit donc d'un amendement de clarification, de précision et de pragmatisme.

: ces amendements visent à proposer le calcul des charges indirectes comme une quote-part des dépenses de fonctionnement de la commune. On risque là d'avoir des résultats aléatoires, alors qu'il sera possible d'ajuster le niveau d'estimation des dépenses, y compris les charges indirectes.

en tenant compte de la jurisprudence abondamment évoquée jusqu'à présent. La crainte du Gouvernement concernant l'intégralité de ces amendements, y compris celui de la commission,

prévu par le Gouvernement visant explicitement à prétendument « responsabiliser les collectivités locales » en mettant à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l'illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe. Par ailleurs, les délibérations relatives à la TEOM n'échappent pas au contrôle de légalité réalisé par les préfectures sur les budgets locaux. De plus, l'État perçoit 3,6 % de la TEOM en contrepartie des frais de dégrèvement. Eu égard à ces deux éléments, je propose de supprimer les alinéas

la coexistence d'une tarification incitative et d'une tarification classique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère, au sein d'une même commune ou d'un même EPCI. Il s'agit de permettre aux collectivités de conduire de vraies expérimentations et aux entreprises prestataires de leur proposer des solutions techniques plus robustes.

Le présent article fixant la nature des charges pouvant être financées par la TEOM, les collectivités ne peuvent plus surfinancer le service et un tel plafonnement devient inutile. Sa suppression permettra de sécuriser l'action des collectivités qui s'engagent dans la TEOM incitative, et ce sans aucun impact sur la fiscalité des ménages. La mesure de plafonnement des recettes de TEOM incitative perçues la première année visait initialement à empêcher les collectivités de profiter du passage en TEOMI pour augmenter les impôts et alimenter ainsi le budget général.

Monsieur Kern, Cet amendement vise à diminuer le montant de la TEOM lorsqu'une entreprise contractualise avec un prestataire privé et qu'elle ne bénéficie pas des services municipaux, à condition que le tri 5 flux ou le tri à la source des biodéchets soit mis en place. d'instaurer un abattement de 40 %, équivalent à la part du ramassage des déchets par les collectivités locales.

Si une collectivité ou un EPCI met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l'unique possibilité de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s'appliquent pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle. La mise en place d'une part incitative de la TEOM peut amoindrir l'effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d'intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d'habitation. C'est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l'autonomie fiscale, cet amendement tend à permettre aux collectivités locales et à leurs groupements de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste et les personnes âgées ou handicapées.

Action coeur de ville ». Cela vient d'être dit, créer une nouvelle taxe n'est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu'efficace pour entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse. En outre, l'absence de différenciation de la taxe sur les surfaces commerciales induit une artificialisation additionnelle par la construction de nouvelles voies routières et de parkings. Cet amendement vise donc à moduler progressivement le taux de la TASCOM selon le lieu d'implantation des grandes surfaces pour le doubler à horizon de 2022 pour les installations hors villes et centres-bourgs et et le réduire de 50 % à horizon de 2022 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de bonus-malus. Il introduit également une majoration additionnelle progressive de 50 à l'horizon de 2022, au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d'établissements concernés par la TASCOM hors villes et centres-bourgs à partir du 1 juin 2019. En outre, dans sa dimension « bonus », cette mesure est de nature à réduire le coût d'exploitation des commerces de villes et de centres-bourgs.

à une majoration inférieure, et de renforcer la progressivité de la TASCOM en fonction de la surface de vente des établissements. Cette évolution de la fiscalité est conforme aux préconisations du rapport du Centre d'analyse stratégique portant sur les aides publiques dommageables à la biodiversité. La mesure est également de nature à renforcer les commerces de proximité, ainsi qu'à faciliter la lutte contre le phénomène de désertification commerciale des petites et moyennes villes, dans une logique cohérente avec les objectifs fixés cadre du plan de revitalisation des centres-villes baptisé « Action coeur de ville ». Enfin, elle incitera à un usage plus économe du foncier périurbain et permettra de lutter efficacement contre l'artificialisation des sols.

Monsieur le rapporteur

Cet amendement vise à étendre l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts de stockage et de logistique destinés, notamment, au e-commerce, l'objectif étant de lutter contre l'artificialisation des terres. La TASCOM doit être un outil de régulation de ce phénomène. Pour rappel, l'implantation d'entrepôts logistiques de grandes surfaces participe largement à l'artificialisation des sols, en particulier dans l'espace périurbain, et constitue un usage en expansion rapide, avec plus de 80 % d'augmentation des surfaces depuis 1999. Il s'agit donc de s'attaquer à la recrudescence des entrepôts de stockage, corrélée à l'augmentation du commerce en ligne et au modèle dit du « dernier kilomètre »- être au plus près des consommateurs pour une livraison plus rapide. Ce type de commerce demande trois fois plus de stockage que la distribution traditionnelle. La modification proposée est tout à fait conforme à la doctrine fiscale, selon laquelle la TASCOM est applicable aux établissements ayant pour activité le commerce de détail, indépendamment de la nature des produits vendus. Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, dont l'importance est réelle pour la préservation de nos sols agricoles et pour la biodiversité.

une taxe sur les ventes de logements HLM. Le produit de cette taxe devait contribuer à la participation des bailleurs sociaux, la Caisse de garantie du logement locatif social,

Toutefois, cette taxe doit s'inscrire dans le cadre du projet gouvernemental de développement des ventes de logements HLM et dans la continuité des mesures votées dans la loi ÉLAN visant à réformer le secteur HLM. C'est pourquoi, dès lors que le nombre de ventes de

inéquitable et économiquement contre-productif dans la mesure où il défavorise les entreprises de transport françaises sans contribuer suffisamment au financement des dépenses d'entretien de la voirie rendues nécessaires par la circulation des véhicules à fort tonnage ». À l'heure où le Gouvernement souhaite supprimer les petites taxes,

Il s'agit de supprimer la taxe pour les collectionneurs de poids lourds, qui ne sont pas très nombreux et roulent très peu.

pour un coût de 40 millions d'euros, ce qui donnera néanmoins plus de lisibilité à la fiscalité française, la contribution annuelle sur les revenus locatifs, le prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, la taxe annuelle sur les médicaments pharmaceutiques vétérinaires et, enfin, les cotisations des entreprises cinématographiques. Je suis saisi

contre les taxes à faible rendement pullulant dans notre système fiscal. Ces taxes sont coûteuses à collecter pour un rendement réduit, voire inexistant. Il peut donc être utile de les supprimer. Toutefois, par le présent sous-amendement, je tiens à attirer l'attention sur deux d'entre elles, qui constituent des ressources du CNC. La première est le prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique. Certes, le rendement de ce prélèvement est très largement symbolique, de l'ordre de 130 000 euros. Pour autant, même en matière fiscale, le symbole est important. Nous pourrions être accusés d'aller à contre-courant d'un mouvement qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et l'exposition de la violence sur les écrans- je pense notamment aux plus jeunes. Il faut cependant reconnaître la pertinence de l'analyse de notre collègue. Aujourd'hui, la pornographie est très majoritairement diffusée sur internet. Peut-être faut-il réfléchir à une évolution de la taxation, mais pensons-y avant de supprimer les dispositifs existants. Les conséquences de la suppression du second ensemble de ne sont pas, pour le coup, symboliques. Il s'agit des cotisations dues par les entreprises de production et de distribution, d'exportation et d'exploitation d'oeuvres cinématographiques. Leur suppression poserait deux types de problèmes. D'une part, si,

Je rappelle que le CNC reçoit environ 680 millions d'euros des trois grandes taxes affectées et prélève un peu plus de 5 % pour son fonctionnement,

D'autre part, la collecte de ces cotisations permet au CNC de contrôler l'ensemble des recettes d'exploitation. Le paiement des cotisations oblige ainsi toute la filière cinématographique à déclarer, auprès du CNC, ses recettes d'exploitation. centre joue, à ce titre, le rôle de tiers de confiance du secteur, en centralisant la totalité des déclarations et en assurant leur suivi. J'espère, mes chers

de trois taxes affectées au budget général de l'État. Ces trois taxes présentent un rendement total d'environ 50 millions d'euros et frappent les mêmes redevables avec une même assiette, mais elles répondent à des règles différentes, notamment pour le calcul de l'impôt et les obligations déclaratives

qui a pour objet d'approfondir la simplification des droits d'enregistrement frappant les actes de la vie des sociétés initiée par l'article 9 du projet de loi de finances dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Son produit est réparti entre communes et EPCI en fonction des dépenses engagées pour l'accueil des gens du voyage. La suppression de cette taxe, malgré la faiblesse de son produit ou la complexité de son recouvrement, se fait sans compensation aux collectivités territoriales

dans sa composante artisanale ainsi que ses spécificités, intrinsèques à l'itinérance qui la caractérise. C'est le seul organisme institutionnalisé représentant les transporteurs fluviaux. Instituée comme le guichet unique de la profession, la CNBA joue le rôle de chambre de métiers pour les bateliers, ce qui confère à ces derniers le double statut d'artisan et de commerçant. L'établissement fonctionne grâce à une taxe parafiscale qui lui est affectée. Financièrement autonome, elle ne bénéficie d'aucune subvention pour charges de service public. La suppression de l'unique représentation institutionnelle de la batellerie se traduira à court et moyen terme par un affaiblissement de la représentation des transporteurs fluviaux artisans, artisans, tant au niveau national qu'européen. Déstructurée, la profession ne serait plus à même de défendre ses intérêts à l'échelle nationale, mais aussi communautaire. Tandis que la batellerie artisanale française connaît actuellement de profondes mutations marquées notamment par des enjeux économiques, réglementaires et environnementaux forts, il est essentiel pour de disposer d'une représentation capable de coordonner l'action de ses entreprises, de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et de contribuer à l'adaptation de la capacité de la flotte. Il apparaît donc que, au lieu de dissoudre la CNBA, il faut au contraire moderniser ses compétences pour lui permettre de servir au mieux les bateliers.

février 2018 la Cour des comptes fait un triple constat : d'abord, la création d'un établissement public administratif en 1982 était justifiée par le caractère administré des relations commerciales dans le transport fluvial de marchandises, mais ce mode de transport a été libéralisé en 2000 ensuite, le statut d'établissement public ne semble plus adapté aux missions assurées par la CNBA et occasionne des modalités de gestion trop lourdes au regard de la taille réduite de l'établissement ; enfin, la gestion de la CNBA nous paraît défaillante- en tout cas, elle est considérée comme telle par la Cour des comptes -, puisque ses ressources, dont la principale d'entre elles est la taxe prélevée sur les bateliers, qui représente 1 500 euros par entreprise et par an, servent principalement à financer son fonctionnement, sans bénéficier suffisamment à la profession.